adopté sous les réserves d’usage. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux

élus locaux, votée à l’unanimité au Sénat en octobre dernier ; moins de six mois plus tard, nous voilà réunis pour examiner le texte établi par une large majorité transpartisane en commission mixte paritaire. Nous pouvons collectivement être fiers du travail accompli. Les violences exercées à l’encontre des élus sont insupportables et nous ne pouvons, à cet égard, que rendre hommage au dévouement et à l’implication des maires qui, sur le terrain, sont plus que jamais les vigies de la République en ces temps difficiles. Si les élus locaux, et singulièrement les maires, doivent bénéficier à tout moment de la protection effective de notre République, celle ci est aujourd’hui largement perfectible. Déposée le 28 mai dernier, peu de temps après la démission de Yannick Morez, alors maire de Saint Brevin les Pins, et avant même que le Gouvernement ne prenne conscience de la nécessité de faire évoluer rapidement les dispositifs en vigueur, la proposition de loi

Fruit d’un travail réalisé en bonne intelligence avec les associations d’élus locaux et les sénateurs de tous les groupes politiques, le texte initial comportait des mesures utiles, largement inspirées de travaux parlementaires antérieurs. Toutes les dispositions initiales ou nouvelles adoptées par le Sénat ont été reprises par l’Assemblée nationale, en commission comme en séance publique. Certaines modifications, sur l’initiative de la rapporteure Violette Spillebout ou de nos collègues députés Thibaut Bazin ou Paul Molac, ont permis d’introduire de nouvelles dispositions particulièrement bienvenues. Je pense en particulier à la disposition visant à conférer le caractère de dépense obligatoire aux dépenses liées à la protection fonctionnelle des élus. De plus, deux dispositions visant à mieux prendre en compte la situation des anciens élus victimes de violences du fait de décisions prises durant leur mandat ont été judicieusement introduites.

allongeant les délais de prescription des personnes dépositaires de l’autorité publique victimes d’injure et de diffamation publiques. Le vote du Sénat avait été unanime – avec votre assentiment, madame la ministre. Les députés se sont opposés à cette évolution,

Il nous faudra impérativement, à l’avenir, renforcer la protection des élus locaux et des personnes dépositaires de l’autorité publique. Ils font face à une multiplication des injures et des faits de diffamation sur les réseaux sociaux, qui prennent une ampleur particulièrement préoccupante. Pour conclure, l’ensemble des dispositions que nous vous présentons aujourd’hui apporteront, j’en suis convaincue, des réponses concrètes et opérationnelles aux difficultés que nos maires rencontrent quotidiennement sur le terrain.

le Sénat, tout comme l’Assemblée nationale, pour le travail fourni sur le sujet de la lutte contre les violences faites aux élus. Nous avons échangé à de très nombreuses reprises

de la lutte contre les violences faites aux élus, au même titre que le plan national de prévention et de lutte contre les violences aux élus. Le phénomène des violences contre les élus est un véritable fléau. S’en prendre à un élu, c’est s’en prendre à la République : il était important

Nous ne pouvons que nous en féliciter collectivement. Cette proposition de loi comporte des avancées législatives majeures, qui viendront compléter les mesures que nous avons prises jusqu’à

Le dispositif repose notamment sur la mise en œuvre d’un « pack sécurité ». Il s’appuie sur la création d’un réseau de plus de 3 400 référents atteintes aux élus » dans toutes les brigades de gendarmerie et dans tous les commissariats, afin que les élus aient un point de contact privilégié pour parler des menaces ou des violences dont ils font l’objet.

ministère de la justice, direction générale des collectivités locales (DGCL). Ce centre a pour objectif de mieux coordonner l’action de toutes les parties prenantes. Il vise notamment à mieux comprendre le phénomène et à examiner les situations individuelles sensibles afin de vérifier la mise en place, au niveau déconcentré, des mesures les plus adaptées pour protéger les élus. Je souhaite que nous ne passions à côté d’aucune situation problématique, et nous devons prendre en charge chacune de ces situations avec la plus grande humanité.

les élus sont confrontés à une violence grandissante dans notre société ; ils sont en première ligne – vous l’avez dit, madame la rapporteure. Les attaques physiques et verbales et le sentiment d’impunité qui découle de ces actes, trop souvent impunis, n’entraînent qu’épuisement chez les élus locaux et les conduisent de plus en plus à des démissions. Ce renoncement, ce désabusement, vous les combattez, nous les combattons. C’est une réponse commune que la République doit apporter pour mieux protéger ses élus. S’il s’intéresse aux sanctions, à la protection et à l’accompagnement des élus, ce texte n’est à nos yeux qu’une première étape. Ce mal qui nous ronge a des racines plus profondes. Encore une fois, je me félicite des travaux que nous menons avec vous sur le statut de l’élu ; ils viendront nourrir la réflexion globale que nous devons mener sur le rapport de notre société à la République et à ses représentants. Le mandat de maire – ce ne sont pas les sénateurs qui me contrediront – est le plus beau mandat. Nous devons le protéger, de même que nous devons protéger tous les élus, qu’ils soient locaux ou nationaux. À ce titre, je voudrais avoir une pensée pour votre collègue, le sénateur Patriat, dont le domicile a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi. Ces actes sont inacceptables, les auteurs doivent être systématiquement et durement punis. C’est la raison qui nous réunit aujourd’hui.

Dans une circulaire conjointe signée par le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux et moi même, que nous avons diffusée à l’été 2023 et qui s’adresse simultanément aux parquets et aux préfets, nous demandons aux procureurs de mettre en place un traitement priorisé des procédures liées aux atteintes aux élus et d’apporter une réponse pénale systématique, ferme et rapide. La circulaire demande que la voie du défèrement soit privilégiée, au regard de la nature des faits et de la personnalité du mis du mis en cause, afin de permettre le prononcé d’une mesure de sûreté, destinée notamment à prévenir toute réitération à l’encontre de la victime.

satisfaisante. Nous devons faire encore mieux et encore plus vite. Ce texte s’inscrit dans une prise de conscience globale, dans une volonté d’action transpartisane. Il vient enrichir le plan national de prévention et de lutte contre les violences aux élus que nous sommes en train de mettre en œuvre, s’appuie pleinement sur votre proposition de loi. Ce plan cherche à agir selon quatre axes : la protection juridique, la sécurité physique des élus, la réponse judiciaire et les relations entre les maires et les parquets. Nous travaillons ainsi à la mise en place d’un dispositif d’aide aux victimes et d’appui psychologique aux élus victimes de violences. Nous trouvons également de nouveaux moyens d’assurer la sécurité physique des élus, notamment en encourageant le déploiement de solutions de vidéosurveillance, qui permettent d’identifier les auteurs et de faire avancer très rapidement les enquêtes. De très nombreux points nécessitent toutefois de modifier la loi, pour renforcer la protection fonctionnelle, améliorer sa prise en charge financière

la voie retenue soulevait de nombreuses inquiétudes. Sur ces sujets, nous devons être capables de trouver les solutions les plus consensuelles possible, et je m’engage à continuer d’y œuvrer avec vous.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

le 21 décembre dernier, à la vue du mot « maire » inscrit sur l’insigne bleu blanc rouge accroché au revers de la veste d’André Mondange, un groupe d’extrême droite a agressé violemment le maire de Péage de Roussillon et sa famille.

Malheureusement, les cas similaires sont nombreux sur tout le territoire français, et je voudrais ici rendre hommage aux très nombreux élus touchés par ce fléau. En 2022, 2 265 plaintes et signalements pour violence verbale ou physique contre des élus ont été recensés par le ministère de l’intérieur,

de mort. La France compte plus de 520 000 élus locaux engagés au quotidien pour défendre les valeurs de la République, dans l’ensemble des 35 000 communes de notre pays. Il est de notre devoir de protéger les représentants de la démocratie locale et d’éviter à la République de se voir ainsi affaiblie,

Si les violences subies par les élus ne sont pas l’unique raison de ce désengagement, nous partageons le constat, mes chers collègues, que ces violences ne peuvent qu’aggraver la chute des vocations. proposition de loi répond à ce besoin en renforçant le volet répressif, afin de mieux protéger nos élus, et en améliorant leur prise en charge lorsqu’ils sont victimes de violences. Toutefois, elle devra aussi s’accompagner d’un réel réinvestissement de l’État dans l’ensemble du territoire français.

La perte d’autonomie fiscale et financière des collectivités affaiblit le pouvoir d’action des élus locaux. Ils sont de plus en plus sollicités, sans pouvoir répondre à tous les besoins de la population, alors qu’ils deviennent l’unique interlocuteur de nombreux citoyens. Il convient donc de protéger les élus dans l’exercice de leur mandat et de veiller en même temps à garantir aux collectivités des moyens d’agir. Si cette proposition de loi et l’accord trouvé sur ce texte répondent à un besoin urgent de sécurité pour nos élus, il nous faudra aussi accepter l’idée que l’échelon communal est essentiel pour l’équilibre de notre République. Nos premiers travaux sur la construction d’un statut de l’élu local de l’élu local sont primordiaux et s’inscrivent dans notre souhait commun de permettre aux élus d’exercer leur mandat dans les meilleures conditions possible. Une réponse répressive ne suffira pas. Nous devons réinvestir tous les territoires de la République, grâce à des services publics fonctionnels et accessibles à tous.

de chacun de ces drames, qui ne sont que les plus médiatisés, l’intégrité physique des élus et la sécurité de leurs proches se sont retrouvés au centre de violences ahurissantes et inacceptables. Au travers des agressions de ces femmes et de ces hommes engagés pour la collectivité, c’est la République qui est attaquée. Aussi, je tiens à saluer la prise de conscience qui a suivi ces tragédies et le travail effectué par notre assemblée,

coûts liés à la protection fonctionnelle des élus municipaux ; elle a également mis en place un dispositif de compensation par l’État des frais occasionnés par cette obligation pour les communes de moins de 3 500 habitants.

Ainsi, l’alignement des peines sur le régime applicable à certains dépositaires de l’autorité publique, l’institution d’une peine de travail d’intérêt général (TIG) en cas d’injure publique ou encore la circonstance aggravante en cas d’atteinte à la vie privée et familiale, instaurés aux premiers articles et à l’article 10 du texte, durcissent la réponse pénale et répondent en cela aux demandes des élus. Les articles 3 à 8 améliorent l’application et le financement de la protection fonctionnelle des élus, qu’ils étendent aux conseillers régionaux et départementaux ainsi qu’aux candidats aux élections locales, en assurant la sécurisation des lieux de réunions en période électorale. Enfin, les articles 11 à 14 visent à renforcer la prise en compte des réalités du mandat par l’appareil judiciaire, contribuant ainsi à une meilleure collaboration du parquet et des services de sécurité de l’État, notamment dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Vous l’aurez compris, mes chers collègues, que l’adoption de ce texte contribuera à une meilleure sécurisation de nos élus locaux et de leurs proches. Notre République démocratique ne peut exister sans le dévouement et les convictions de tous ceux qui œuvrent chaque jour à sa préservation, à son fonctionnement et à son rayonnement. Il est de notre devoir de leur assurer protection, ainsi qu’à leurs proches. Conscient de cet enjeu crucial, le groupe RDSE votera à l’unanimité le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire. La parole

renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, élus qui font face, ici comme en outre mer, à une hausse inquiétante des violences à leur encontre. À mon tour, j’ai une pensée toute particulière pour le président Patriat. La commission mixte paritaire s’est réunie le 27 février dernier ; elle est parvenue à un accord, dans l’intérêt de nos élus locaux. Le présent texte vise un objectif important et consensuel. Dans cet esprit, il a fait l’objet d’un travail de coconstruction entre les deux assemblées et le Gouvernement. tout d’abord, une traduction dans la loi d’une partie des mesures du plan national de prévention et de lutte contre les violences aux élus présenté par le Gouvernement en juillet 2023. Le texte comportait initialement des mesures utiles, auxquelles la navette parlementaire a apporté un certain nombre d’améliorations. Nous pouvons nous réjouir que l’Assemblée nationale en ait préservé les grands équilibres et qu’elle ait conservé les apports du Sénat.

une peine de travail d’intérêt général en cas d’injure publique à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou de certains élus sera créée, de même qu’une circonstance aggravante en cas de harcèlement. texte prévoit également des mesures pour améliorer la prise en charge des élus locaux victimes de violences. L’octroi de la protection fonctionnelle sera automatique les maires et les adjoints, ou anciens maires et adjoints, victimes de violences, de menaces ou d’outrages qui en feront la demande.

Enfin, même si le Sénat n’en est pas friand, plusieurs demandes de rapport ont été introduites dans le texte. Elles portent sur l’opportunité d’élargir la protection fonctionnelle à l’ensemble des élus locaux, y compris à ceux qui n’exercent pas de fonctions exécutives sur les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et sur leurs résultats, en vue de disposer de statistiques plus précises concernant les élus locaux ; enfin, sur le coût, pour les communes, de l’obligation de souscrire un contrat d’assurance couvrant les frais liés à la protection fonctionnelle. Il restait néanmoins quelques points de divergence qui ont fait l’objet de compromis, à l’exception de l’article 2 , introduit au Sénat, qui prévoyait l’allongement des délais de prescription des délits d’injure et de diffamation publiques, pour les porter de trois mois à un an. L’Assemblée nationale souhaitait, quant à elle, en restreindre l’application aux élus locaux. Outre l’objectif de favoriser la liberté d’expression, le choix d’enserrer les possibilités d’action judiciaire contre les délits de presse dans des délais restreints était justifié par le caractère éphémère de la presse papier et la rapide disparition du support de l’infraction, justification qui ne tient plus avec avec l’évolution des techniques de communication. Avec François Pillet, nous avions déjà réfléchi sur ce sujet, en juillet 2016, dans un rapport d’information intitulé.

et à la citoyenneté, des amendements visant à adapter le régime de la prescription des délits de presse aux spécificités d’internet, qui rendent difficilement identifiable l’auteur des faits et permettent à des messages délictueux de perdurer dans l’espace public. C’est pourquoi, à titre personnel, je pense que la version retenue par le Sénat allait dans le bon sens et prenait en compte cette évolution impérative de notre droit aux nouvelles technologies des moyens de communication. Il est regrettable que nos collègues députés ne l’aient pas voté en termes identiques. Pour autant, et malgré ce regret, l’unanimité ayant été acquise au Sénat en première lecture pour la protection de nos élus, le groupe RDPI confirmera son vote en faveur de son adoption, dans les mêmes conditions.

se banalisent, tous les corps de la société sont touchés : les journalistes, les enseignants, les sapeurs pompiers, les médecins, et aussi les élus. Chaque fois qu’un élu est attaqué, que ce soit verbalement ou physiquement, nous témoignons unanimement de notre soutien et de notre solidarité à l’égard de la victime. Chaque fois, nous clamons toutes et tous notre indignation, sans que les sources de cette violence se tarissent, sans que notre législation arrive à l’endiguer, malgré de nombreuses initiatives parlementaires. Nous le constatons toutes et tous dans nos territoires, qu’ils soient ruraux, urbains ou périurbains : face à une tension généralisée, ce sont désormais les maires et les élus municipaux qui sont en première ligne. Mobilisés au quotidien, ils sont les premiers à faire face au mécontentement de nos concitoyens. ce mécontentement se transforme parfois, et de plus en plus souvent, en violence physique ou verbale, dont les élus locaux sont alors les premières victimes. Il devient donc impératif que notre droit évolue et se fasse plus protecteur à leur égard.

l’octroi automatique de la protection fonctionnelle aux maires, aux élus municipaux, aux suppléants ou aux personnes ayant reçu une délégation, lorsque ces derniers sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages, ou encore le dépaysement des affaires mettant en cause un maire ou un adjoint dans l’exercice de leur mandat. Ces mesures sont de bon sens et vont dans le bon sens. Elles seront de nature à protéger nos élus par un arsenal pénal renforcé, à améliorer leur accompagnement et leur prise en charge lorsqu’ils sont victimes de violence physique ou verbale, tout en leur assurant un traitement judiciaire équitable et raisonné lorsque cela est nécessaire. Nous regrettons cependant que nos propositions visant à étendre la protection fonctionnelle à tous les élus, notamment ceux d’opposition, n’aient pas été adoptées. Un rapport en la matière est bienvenu, mais largement insuffisant. Pourquoi attendre, alors que le bon sens dicte De la même manière, les revirements de l’Assemblée nationale sur l’allongement des délais de prescription des délits d’injure et de diffamation publique commis à l’encontre des élus restent, à ce jour, problématiques, dans la mesure

Ces regrets étant énoncés, formons le vœu que ce texte soit utile pour celles et ceux qui incarnent la République partout en France. Grâce à cette proposition de loi, nous adressons un message aux élus de l’Hexagone et des territoires ultramarins,

un sujet qui traverse notre société et touche de plein fouet l’ensemble des élus de la République. Pour ce faire, nous avions essayé d’apporter des réponses

même de souligner la réactivité du Sénat sur l’ensemble de ces sujets, puisque, dès 2019, certains collègues l’ont rappelé, à la suite du décès du maire de Signes Jean Mathieu Michel, la commission des lois s’était fixé comme objectif prioritaire de travailler sur le sujet des violences auxquelles sont confrontées les élus, en y apportant des réponses très concrètes. Nous l’avons dit, notamment, dans le cadre du texte Engagement et proximité. Nous avons poursuivi la réflexion en faisant écho

enthousiasme que le groupe Les Républicains votera ce texte, qui appelle bien sûr des réponses complémentaires. La parole Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voilà réunis pour la conclusion du chemin parlementaire d’un texte particulièrement important. Comme vous, j’ai pu mesurer, lors de mes multiples rencontres avec les élus locaux, comme dans mon expérience au sein de ma commune, la problématique lancinante et intolérable de l’agressivité dont les élus peuvent faire l’objet. Dans ce domaine, quelques chiffres doivent être rappelés – et ils l’ont déjà été. Notre assemblée a produit un travail de qualité pour évaluer et circonscrire ce phénomène délétère. Depuis la crise sanitaire de 2018 et les émeutes de l’été dernier, qui ont ravagé de trop nombreuses communes, les élus locaux font face à une flambée de violence endémique à leur égard. en 2019 par notre collègue Philippe Bas, 92 % des élus interrogés avaient enduré des incivilités, des injures ou même des agressions physiques. Selon le ministère de l’intérieur, en 2023, 2 300 atteintes aux élus ont été enregistrées, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. Nous sommes particulièrement sensibles à la question de la protection des élus, car nombre de mes collègues députés, conseillers régionaux, départementaux ou municipaux ont déjà fait les frais de cet ensauvagement, qui dégrade sans cesse la vie d’élu local et empêche de plus en plus nos concitoyens de s’engager dans ces beaux mandats, au service de nos territoires. Bien évidemment, toute violence verbale ou physique contre des représentants du peuple, quelle que soit leur appartenance politique, est insupportable. Nous déplorons que l’œcuménisme ne soit pas toujours partagé en la matière. Le texte qui nous est ainsi présenté apporte des mesures utiles à la protection de nos élus. L’élargissement de la protection fonctionnelle octroyée aux élus et l’inscription en dépense obligatoire de la protection fonctionnelle constituent des avancées bienvenues. Néanmoins, à l’instar de notre collègue Catherine

Nous nous félicitons que des mesures déterminantes aient été votées pour protéger les candidats aux élections locales. De même, le renforcement des sanctions pénales contre les auteurs de violences à l’encontre de nos élus va dans le bon sens. Nous devons, dans ce domaine comme dans d’autres, appliquer le principe de la tolérance zéro. Sitôt ce texte adopté, il nous faudra rester vigilants quant à la publication des décrets d’application, ainsi qu’à la traduction pénale des mesures que nous aurons adoptées. Madame la ministre, la sécurité des élus locaux est un principe non négociable. Nous approchons, lentement mais sûrement, des élections municipales de 2026. avec ses 500 000 élus locaux, d’une armature démocratique à nulle autre pareille. L’insécurité et l’incivilité latentes de notre société ne peuvent plus dégrader la vie, déjà bien difficile, de nos élus locaux, garants et défenseurs de notre identité républicaine. Ce texte ne constitue pas la fin de notre travail, mais bien l’amorce de notre réarmement pénal contre l’insécurité touchant nos élus, comme tous les Français. À ce titre, vous nous trouverez toujours au rendez vous de la sérénité et de la sécurité de nos compatriotes, quels qu’ils soient. La parole est à M. Vincent Louault, pour le groupe

permettant d’améliorer le mandat des élus locaux grâce à un grand nombre de dispositions concrètes et bienvenues. Aujourd’hui, c’est le volet sécuritaire qui nous réunit, sujet ô combien important ! Cette proposition de loi est attendue de très longue date. En cette période de crise de l’engagement, il était nécessaire de proposer de nouvelles solutions pour protéger les élus dans l’exercice de leur mandat. Ce texte a été malheureusement rendu nécessaire par les récents drames qui se sont succédé ces derniers mois et la hausse des violences, injures et incivilités envers les élus locaux. Pis, ces violences intolérables sont en hausse, comme nous le martelons régulièrement au Sénat. Selon un récent rapport du ministère de l’intérieur, plus de 2 000 plaintes ou signalements ont été recensés en 2022, soit une augmentation de 32 % en un an. La parole s’est aussi libérée. Dès 2020, le garde des sceaux et le ministre de l’intérieur sont montés au créneau avec, en la matière, des consignes fortes et courageuses, renforcées par votre circulaire, madame la ministre. En plein contexte de crise démocratique, il faut couper court à cette vague de violences. Je souhaite saluer les auteurs de ce texte et ses rapporteurs. Nous nous sommes félicités en octobre dernier d’avoir adopté ce texte, avant qu’il ne soit examiné par l’Assemblée nationale, le 7 février 2024. Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir, puisque la commission mixte paritaire est parvenue à une rédaction commune de l’ensemble des dispositions restant en discussion. Nous regrettons le rejet de l’allongement des délais de prescription en cas d’injure et de diffamation publiques envers des personnes dépositaires de l’autorité publique. C’était pourtant une bonne avancée. Nous espérons que le Gouvernement pourra s’en emparer. Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire reprend largement les apports du Sénat. Je pense, par exemple, à la mesure permettant la répression pénale de toute atteinte à la vie privée des candidats à un mandat électif. Il s’agit d’une bonne disposition. Saluons ce travail collectif, qui permet d’aboutir à un texte concret, efficace et ambitieux. Il aidera utilement nos élus dans l’exercice de leurs fonctions. Madame la ministre, il s’agit de poursuivre les efforts en faveur de la protection des élus, qui œuvrent au quotidien auprès de leurs administrés, ne ménageant ni leur temps ni leur peine. Par ce texte, nous reconnaissons et saluons leur engagement de tous les instants au service de leur territoire. Nos élus peuvent compter sur notre entière mobilisation à leurs côtés. Cette proposition de loi en est une preuve supplémentaire. Il s’agit désormais de les accompagner au plus près de leur mandat, en s’assurant que l’ensemble des services judiciaires, administratifs et étatiques mettent en œuvre toutes les mesures pour les protéger. C’est simple, si nous voulons dissuader les fauteurs de troubles et de violences, il faut punir plus fort et systématiquement. Nos élus attendent de la fermeté, et cette loi le permettra. Mes chers collègues, vous l’aurez compris, notre groupe soutient avec force ce texte si important pour nos élus locaux. La parole

je tiens tout d’abord à saluer tous les élus victimes d’agression. J’ai une pensée particulière pour l’ancien maire de Signes, Jean Mathieu Michel, mortellement blessé en août 2019 par le conducteur d’une camionnette qu’il voulait verbaliser pour avoir jeté des gravats sur le bord de la route.

Le résultat est là : en quelques articles sont clairement posés l’aggravation des peines en cas d’agression contre un élu ou contre un ancien élu, ce qui permet de sanctionner des personnes malveillantes attendant attendant la fin du mandat d’un élu pour agir violemment contre lui, la protection des candidats à un mandat électif, l’élargissement du bénéfice de la protection fonctionnelle, et le droit à l’assurance pour les permanences des élus et des candidats à un mandat. Aujourd’hui, nous allons donc apporter une réponse circonscrite à des actes de violence ayant pris de l’ampleur depuis des années. Si j’use du mot « circonscrit », c’est à bon escient : il ne s’agit nullement de diminuer la qualité du travail qui a été réalisé.

Ces textes contribuent à améliorer le quotidien des 500 000 élus que compte la France. Mais suffiront ils à répondre au malaise qui s’empare de nombre de nos collègues

En mars 2020, lors des élections municipales, 106 communes s’étaient retrouvées sans candidat déclaré. En 2014, les communes sans prétendant à la fonction de maire étaient au nombre de 62, soit une hausse de 70 Ce désarroi a des origines complexes. Il est ainsi possible d’évoquer une forme de repli sur soi ou sur son proche entourage, une peur de l’engagement, qui entraîne trop d’obligations, ou une moindre appétence pour la chose publique due à la dégradation du débat public.

Être élu, selon notre conception de la démocratie, c’est avant tout un engagement volontaire et personnel. Mais peut on imaginer qu’être élu devienne un métier qui nécessiterait un diplôme ? Il existe, depuis des années, des formations pour devenir collaborateur d’élu. Peut être faudrait il en créer une pour être élu ? Il y a aujourd’hui une telle suspicion à l’égard de la politique et des élus, considérés par la plupart des Français comme des privilégiés, qu’élus, avons peut être peur d’aborder ces questions. Ces pistes de réflexion sont ouvertes à tous. Pour revenir au présent texte, comme nous l’avons dit en commission des lois, toutes les évolutions législatives que nous pouvons adopter doivent nécessairement s’accompagner d’un changement de culture des acteurs judiciaires et étatiques, lesquels ne peuvent plus rester passifs face à cette violence. Enfin, je tiens

Notre chambre, dans son ensemble et sa diversité, restera toujours attentive aux problématiques de nos élus et de nos institutions locales. Ses nombreux travaux montrent et démontrent le besoin d’un renouveau de la démocratie locale, à laquelle nous sommes très attachés. Notre démocratie doit accompagner et susciter la volonté d’engagement citoyen dans les projets et actions de transformation et de transition, au cœur de nos territoires. La crise de confiance et la crise de l’engagement sont profondément liées. Le besoin de redonner aux élus locaux leur pouvoir d’agir dans de bonnes conditions, le besoin de conforter leur rôle essentiel de proximité auprès de nos concitoyens, la nécessité de revitaliser l’engagement citoyen, passent aussi par leur protection. À ce titre, les écologistes ont toujours activement soutenu les réflexions sur le sujet et proposé des solutions permettant de désamorcer le niveau de tension existant entre élus et citoyens, qui a parfois entraîné des dérives violentes inacceptables.

Notre groupe soutient l’action des élus locaux et s’associe à l’ensemble des propositions qui pourraient leur permettre une plus grande protection, un meilleur accompagnement dans leur engagement. Souvent non indemnisée, la conciliation avec leur vie professionnelle et personnelle peut être un frein à leur implication. Nous nous associons à la demande d’un véritable statut de l’élu plus protecteur et du développement de moyens concrets d’accompagnement pour améliorer la parité et la diversité des profils. Cette proposition de loi ne résoudra pas ces crises.

Les périodes de campagne étant propices au déclenchement de violences, il est bienvenu que ce texte permette aux candidats déclarés d’être couverts par le mécanisme de protection fonctionnelle. Enfin, nous ne pouvons que soutenir les dispositifs liés à la facilitation des relations avec les acteurs judiciaires et saluer l’équilibre nécessaire trouvé, en dépaysant d’office les affaires dont l’élu serait le mis en cause. De manière générale, nous soutenons les mesures inscrites dans cette proposition de loi. Pour autant, nous sommes très attentifs à ce que ce renforcement de la protection des élus ne puisse être perçu comme un ensemble de mesures inéquitables, accroissant ainsi le fossé entre élus et citoyens. La hausse des violences envers les élus doit toutes et tous nous alerter et nous faire réagir, en tant que parlementaires, bien sûr, mais aussi et surtout en tant que citoyens. Notre message est clair : quelles que soient leurs formes, les violences à l’égard des élus ne sont pas tolérables dans notre société et doivent être condamnées.

et une meilleure utilisation des moyens en ce sens. Oui, il est essentiel d’encourager et d’accompagner les dépôts de plainte pour violences envers les élus, car il est essentiel d’encourager et d’accompagner les dépôts de plainte pour l’ensemble des violences, notamment les violences au travail ou les violences sexistes et sexuelles. Nous devons continuer de nous interroger sur le sentiment d’être perdu dans le parcours du combattant de la judiciarisation des actes subis par les victimes. Mais nous ne sommes pas dupes Ces violences contre les élus, aussi inacceptables et injustifiables soient elles, s’inscrivent dans la perception d’un fossé entre le politique et le citoyen, la fin de la croyance d’une gouvernance pour l’intérêt commun, le sentiment accru d’une déconnexion entre la volonté citoyenne et l’action du politique, entre la vie au quotidien et notre capacité à la modifier. La montée des violences trouvera aussi une réponse au travers d’un développement plus large de la démocratie locale. Attelons nous à imaginer et initier des référendums citoyens, des budgets citoyens, des implications citoyennes bien en amont des décisions. Pour toutes ces raisons, et conscient des risques et limites de cette proposition de loi, notre groupe votera ce texte.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023 389 du 24 mai 2023 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Polynésie française

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi de ratification de l’ordonnance du 24 mai 2023 s’inscrit dans une démarche de clarification et d’harmonisation, pour un droit plus lisible

Pendant longtemps, le droit domanial applicable à la Polynésie est resté illisible en raison des nombreux régimes applicables et des différentes catégories de domaines. Depuis 1977, la Polynésie française détient la propriété de son domaine, à la suite du transfert par l’État de la totalité de son domaine public maritime à cette collectivité, à l’exception notable des zones dédiées à l’exercice de sa souveraineté, comme celles qu’utilise la marine nationale. Bien qu’ils jouissent d’une grande autonomie en matière de gestion domaniale, l’État et ses institutions publiques conservent un important patrimoine public, incluant des infrastructures telles que les aérodromes, tribunaux, ports ou écoles, ainsi qu’un domaine privé. cours du précédent quinquennat, le Parlement a voté la loi organique du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, et ce afin de simplifier le droit applicable. Cette loi a eu pour effet d’attribuer à l’État la faculté d’étendre les règles applicables à son domaine privé et à celui de ses établissements publics, tout en soumettant les dispositions législatives et réglementaires correspondantes au régime de l’applicabilité de plein droit. Elle a en outre permis d’étendre le régime d’applicabilité de plein droit aux dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine public des établissements publics de l’État, alignant ainsi le régime d’applicabilité de ces dispositions sur celui qui prévalait pour le domaine public de l’État. Ainsi, depuis 2019, les règles relatives aux domaines public et privé de l’État et de ses établissements publics sont applicables de plein droit en Polynésie française. En somme, en cohérence avec ce qui existait déjà dans les autres collectivités d’outre mer, le présent projet de loi prévoit d’harmoniser les règles applicables et de donner à l’État une compétence en matière d’établissement des règles relatives à son domaine privé et aux domaines privé et public de ses établissements publics en Polynésie française. Cette évolution positive méritait d’être mise en œuvre, puisque le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) n’avait pas été mis en cohérence avec ces nouvelles dispositions. Or nous devons à la Polynésie et à nos collectivités d’outre mer un droit pleinement applicable et de qualité. Je sais que vous y êtes très attaché,

afin de rendre plus lisible l’application du droit domanial dans les collectivités concernées. Les règles relatives au domaine privé de l’État en Polynésie française n’ont cependant pas pu entrer dans le champ de cet exercice de codification, le Conseil d’État ayant rendu un avis, le 15 septembre 2016, aux termes duquel a été retenue une interprétation stricte de la compétence de l’État sur son seul domaine public

Elle permet ainsi de compléter la partie législative de ce code consacrée à l’outre mer en renforçant, tant pour les praticiens que pour les usagers, la cohérence et l’intelligibilité des règles de droit domanial applicables en Polynésie française. L’ordonnance est prise sur le fondement de l’article 74 1 de la Constitution, qui confère au Gouvernement une habilitation permanente pour étendre, par ordonnances, dans les collectivités régies par l’article 74 et en Nouvelle Calédonie, les dispositions législatives en vigueur en métropole dans les matières relevant de la compétence de l’État. Si cette ordonnance donne davantage de lisibilité au droit domanial en Polynésie française, elle ne remet aucunement en cause – j’y ai été très attentif – les compétences de la collectivité. Je veux par ailleurs rassurer : je sais que cette ordonnance a pu susciter des interrogations chez certains élus polynésiens, mais je sais aussi que le travail du sénateur Teva Rohfritsch et de sa collègue Lana Tetuanui… ont permis de lever ces doutes. J’en profite pour saluer le travail de concertation et le dialogue entre parlementaires et élus locaux. C’est l’exemple même de la relation de confiance qui doit se nouer pour œuvrer le plus efficacement possible au service de tous les territoires. Je veux également souligner le travail de consultation qui a été mené et je note que l’assemblée de la Polynésie française avait émis un avis favorable sur la loi organique de 2019. Je sais que le dialogue se poursuivra notamment avec la ministre déléguée chargée des outre mer, Marie Guévenoux, qui est actuellement en déplacement en Guyane et que je salue.

prise sur le fondement de l’article 74 1 de la Constitution, l’ordonnance du 24 mai 2023, qui est soumise à la ratification du Sénat, tend à compléter le livre du code général de la propriété des personnes publiques consacré à la Polynésie française. Considérant cette ordonnance comme un facteur d’amélioration de la cohérence et de la lisibilité des règles de droit domanial applicables en Polynésie française, la commission des lois a approuvé sa ratification sans modification.

la multiplicité des régimes applicables et des catégories de domaine rendait en effet peu lisible le droit domanial applicable sur ce territoire. Vous le savez, l’une des spécificités du cadre juridique de la Polynésie française réside dans l’entrecroisement de différents niveaux de compétences normatives. La collectivité dispose d’une compétence normative de principe, tandis que l’État ne peut agir qu’au sein d’un périmètre de compétences qui lui est dévolu par la loi statutaire de 2004. À À cela s’ajoute la coexistence de différentes catégories de domaines. Depuis 1977, la Polynésie française est propriétaire de son propre domaine, auquel l’État a transféré l’entièreté de son domaine public maritime, à l’exception – il est bon de le noter – des dépendances affectées à l’exercice de sa souveraineté, comme celles de la marine nationale. Dans cette collectivité d’outre mer particulièrement autonome en matière domaniale, l’État et ses établissements publics conservent néanmoins la propriété d’un vaste domaine public, qui comprend des aérodromes, des palais de justice, des ports ou des écoles, et d’un domaine privé. Jusqu’en 2019, seul le domaine public de l’État figurait parmi les compétences reconnues aux autorités étatiques par le statut de 2004., l’État n’était pas compétent pour établir les règles relatives à son domaine privé. Cette répartition des compétences était singulière, notamment en comparaison des autres collectivités d’outre mer. À la lumière des auditions que j’ai conduites, elle semble davantage relever d’une omission que d’un choix délibéré. Il en résultait une insécurité, si ce n’est un vide juridique. En effet, bien qu’ayant la compétence théorique pour légiférer sur le domaine privé de l’État, la Polynésie française n’en a jamais fait usage. Dès lors, le domaine privé de l’État se trouvait, en pratique, régi par l’ancien code du domaine de l’État, qui avait été maintenu en vigueur à titre dérogatoire. Cette fragmentation normative a été naturellement préjudiciable à l’intelligibilité, mais également à l’évolution des normes. Comme le relevait le Conseil d’État en 2016, le législateur ordinaire demeurait en effet incompétent pour modifier une disposition touchant au domaine privé de l’État en Polynésie française. Face à ce insatisfaisant, la loi organique du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française a permis de faire un premier pas vers la résolution de cette situation. Elle a ainsi étendu expressément la compétence de l’État en Polynésie française à son domaine privé et aux domaines public et privé de ses établissements publics. Par souci de simplification et de lisibilité, le régime de l’applicabilité de plein droit a été élargi, sur l’initiative du Sénat, au domaine de l’État et de ses établissements publics.

les règles applicables, avec ou sans adaptations, et celles qui ne sont expressément pas étendues. L’ordonnance, que le présent projet de loi tend à ratifier, opère donc cette actualisation quatre ans après. la commission des lois tient à déplorer les lenteurs de la réforme, au regard des enjeux particulièrement prégnants de lisibilité du droit en Polynésie.

Au delà de son aspect très technique, cette ordonnance est emblématique des difficultés juridiques auxquelles sont confrontées les collectivités d’outre mer

à la nécessité de veiller à ce que cet objectif de clarté ne fasse pas fi des spécificités locales et ne conduise pas à omettre toute adaptation et toute prise en compte du statut particulier de la collectivité.

en supprimant par exemple la mention de codes inapplicables en Polynésie ou encore des éléments qui n’ont pas d’équivalent local, comme les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural Le travail le plus important réside finalement dans l’identification des dispositions relevant de la compétence de la Polynésie française. Pour des motifs historiques et politiques, le statut de 2004 réserve en effet à la Polynésie française une compétence exclusive pour acquérir certains biens. Ainsi, la Polynésie française dispose d’un droit de préemption immobilier de même, elle est compétente en ce qui concerne les biens vacants et sans maître ou ceux des personnes qui décèdent sans héritier. Dès lors, l’ordonnance exclut expressément

En tant que rapporteur, je me suis attaché, au cours des travaux préparatoires de la commission, à recueillir l’avis et les observations des représentants polynésiens, le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, le SPCPF, le président de l’assemblée de la Polynésie française et notre collègue Lana Tetuanui. Sans préempter le débat que nous ne manquerons pas d’avoir dans quelques instants, je vous assure avoir accordé la plus grande considération aux réserves formulées par les représentants de la Polynésie française. Toutefois, au terme d’une analyse juridique approfondie, la commission est parvenue à la conclusion que cette ordonnance traduisait fidèlement les principes fixés par la loi organique de 2019, sans empiéter sur les compétences de la Polynésie française. Ainsi, en matière d’acquisition des biens culturels maritimes, l’ordonnance

notre collègue Agnès Canayer ait été déclaré irrecevable, tant son dispositif semblait apporter une réponse attendue à la problématique de l’entretien des chemins privés ruraux en Polynésie. Sensible à ces enjeux, je souhaite qu’un prochain véhicule législatif nous permette d’obtenir des avancées en la matière. En somme, la commission des lois a considéré que le présent projet de loi permettait de clarifier et de mettre en cohérence, avec du retard, mais une certaine prudence, le droit domanial de l’État en Polynésie française. Au bénéfice de ces observations, la commission vous invite, mes chers collègues, à adopter ce projet de loi de ratification sans modification. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous penchons de nouveau aujourd’hui sur les principes fixés par la loi organique du 5 juillet 2019 relative à la répartition des compétences et au régime d’applicabilité du droit domanial en Polynésie française. Cette fois ci, il est question de l’ordonnance du 24 mai 2023 qui consolide les principes émis par la loi organique en modifiant le code général de la propriété des personnes publiques. Avant toute chose, je tiens à saluer le travail dense, riche et efficace du Parlement qui a scellé, par la loi organique de 2019, un pacte de confiance entre l’Hexagone et les collectivités d’outre mer.

Ces caractéristiques appellent naturellement à la mise en place d’un régime juridique exigeant, qui permette aux usagers de mieux s’en prévaloir. Ce texte met donc fin au régime de spécialité législative qui prévalait pour l’application des dispositions relatives au domaine public des établissements de l’État. Il aligne enfin le régime polynésien sur celui de l’applicabilité de plein droit pour ce qui relève du domaine public de l’État. Pour ce territoire, qui s’étend sur une superficie comparable à celle de l’Europe, une telle clarification était nécessaire.

Avant d’être une simple propriété foncière, il est avant tout un symbole affectif, social et culturel. Pour concilier ces exigences culturelles avec les spécificités de nous appelons le Gouvernement à se saisir de nouveau du projet de codification du régime de la propriété publique en Polynésie, abandonné en 2011. Le groupe RDSE s’est toujours prononcé en faveur de tels projets de codification.

est marqué du sceau de la clarification et de la cohérence. Je salue l’excellent travail de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, rapporteur de la commission des lois, qui s’est beaucoup impliqué sur ce texte. Avant 2019, de multiples régimes applicables et différentes catégories de domaines rendaient le droit domanial applicable à la Polynésie française illisible. Le Parlement a voté la loi organique du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française pour remédier à cette Ce texte harmonise les règles applicables aux collectivités d’outre mer et délègue à l’État la compétence en matière d’établissement des règles relatives à son domaine privé et aux domaines privé et public de ses établissements publics en Polynésie française, comme c’était déjà le cas dans toutes les autres toutes les autres collectivités d’outre mer et en Nouvelle Calédonie. Cette évolution, pour positive qu’elle soit, restait incomplète en l’absence de mise en cohérence du code général de la propriété des personnes publiques. Ce sera chose faite avec la ratification de l’ordonnance du 24 mai 2023, qui intervient plus de quatre ans après la promulgation de la loi organique de 2019.

récemment, cette ordonnance a pu susciter quelques interrogations parmi les élus polynésiens, notamment concernant l’appréhension par l’État de la notion de « biens culturels maritimes » situés dans son domaine public maritime. Je souhaite remercier mon collègue Teva Rohfritsch, sénateur de la Polynésie française, qui a travaillé sur ce texte au sein de notre groupe RDPI. Il a tenu à clarifier cette disposition précise auprès de l’assemblée de la Polynésie française qui l’avait interpellé. Je salue également notre collègue Lana Tetuanui sur ce dossier. Tous deux ont réalisé un travail remarquable dans l’intérêt de la Polynésie française.

la zone maritime polynésienne relevant par ailleurs quasi exclusivement de la Polynésie française. Je

de proposer des mesures adaptées à cette géographie de l’immense océan Pacifique, au bénéfice de nos collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et des 550 000 citoyens français qui y résident. toutes ces raisons et avec en tête l’intérêt premier de nos concitoyens de la Polynésie française, le groupe RDPI votera ce texte. La parole

modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Polynésie française. Cette évolution concerne l’utilisation des biens appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et aux organismes publics.

La loi organique de 2019 a permis de clarifier et de préciser les précédentes législations. Ainsi, en accord avec les élus du territoire polynésien, le Gouvernement a élaboré

positif métropolitain et le droit spécifique à la Polynésie française quant à la gestion des biens publics. L’objectif est tout simplement d’améliorer la lisibilité de la répartition des compétences et le régime d’applicabilité du droit domanial en Polynésie française.

Il était donc essentiel de mettre fin aux incertitudes qui entouraient les compétences de l’État et qui avaient pu freiner certaines initiatives

code énonce désormais que les dispositions du code « sont applicables de plein droit en Polynésie française au domaine public et privé de l’État et de ses établissements publics ». Cette modification met fin à toute ambiguïté.

le projet de loi que nous soumet aujourd’hui le Gouvernement s’inscrit dans la continuité des travaux antérieurs du Parlement relatifs à la Polynésie française, en particulier des ajustements au statut de cette collectivité opérés par une loi organique de 2019, dont le rapporteur, au Sénat, était notre collègue Mathieu Darnaud. L’ordonnance qu’il nous est proposé de ratifier concerne la question juridiquement complexe du domaine public de l’État. Cette thématique acquiert une acuité particulière dans les collectivités françaises du Pacifique, sujettes à des règles souvent fortement dérogatoires au droit commun. ainsi de la Polynésie française, territoire doté d’un immense domaine maritime, dont l’autonomie est régie par l’article 74 de la Constitution. L’actuelle répartition du domaine public fut historiquement structurée par un transfert graduel, à partir de 1977, de tronçons du domaine public de l’État à la collectivité polynésienne. La cohabitation des domaines y fut ensuite consacrée par la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dont l’article 46 prévoit l’exercice par l’État, la Polynésie et les communes de leurs droits de propriété sur leurs domaines respectifs. Toutefois, le droit applicable à la domanialité de l’État en Polynésie n’était pas dénué d’ambiguïtés.

Or la Polynésie française dispose de la compétence par principe sur son territoire ; cette omission revenait donc implicitement à laisser la compétence relative à l’encadrement du domaine privé de l’État à la collectivité, contrairement à ce qui existe dans d’autres collectivités ultramarines. Bien que la Polynésie n’en ait pas fait usage, cet état du droit a engendré une complexité inutile et endommagé la sécurité juridique du domaine privé de l’État et de ses établissements publics. En 2019, la loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française a utilement entamé le travail de correction de ce qui s’apparentait clairement à une anomalie et à un oubli. L’applicabilité de plein droit des dispositions nationales relatives aux deux domaines de l’État, public et privé, est donc formellement la norme dans ce territoire depuis cinq ans. Cette modification de la loi organique relative à la Polynésie nécessitait cependant une répercussion au niveau de la loi ordinaire, en particulier au livre VI de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques. Tel est l’objet de l’ordonnance du 24 mai 2023, que l’on nous demande aujourd’hui Je ne reviens pas sur le détail, souvent technique, du contenu de l’ordonnance, dont il suffit de dire qu’elle tire les conséquences de la loi organique et procède à un certain nombre d’adaptations, clarifications et de simplifications rédactionnelles du code, qui amélioreront la lisibilité du droit. À cette occasion, je salue le travail d’analyse accompli par notre rapporteur Thani Mohamed Soilihi, notamment sur la question du domaine public maritime en Polynésie. Enfin,

La loi organique de 2019, qui a modifié le statut de la Polynésie française, a comblé une lacune en mentionnant explicitement la compétence de l’État dans son domaine privé et a étendu le régime applicable de plein droit à toutes les dispositions relatives aux domaines public et privé de l’État.

Parce qu’il est urgent et nécessaire d’améliorer la lisibilité du droit applicable en Polynésie française, le groupe Les Indépendants votera pour la ratification de cette ordonnance. La

Conformément à l’article 74 1 de la Constitution, le Sénat est appelé à examiner, sous peine de caducité, le projet de loi ratifiant l’ordonnance modifiant

ordonnance reprend essentiellement des dispositifs existant en métropole, au bénéfice de la gestion domaniale de l’État. Son esprit est celui d’une meilleure lisibilité du droit. À l’origine, en vertu du partage des compétences entre l’État et la Polynésie, il appartenait à la collectivité d’outre mer de fixer les règles relatives au domaine privé de toutes ses collectivités publiques. L’État a ensuite a ensuite préféré reprendre cette compétence. Cependant, pour que les dispositions législatives relatives au domaine privé de l’État soient applicables, encore fallait il que le texte normatif soit étendu par une mention d’applicabilité.

En effet, le deuxième alinéa de son article 2 prévoit de ne pas étendre à la Polynésie les articles relatifs à certaines modalités d’acquisition

Néanmoins, monsieur le ministre, le dernier alinéa de l’article 2, qui introduit l’acquisition de biens culturels maritimes par l’État, en tant qu’ils sont situés dans son domaine public maritime, appelle une certaine réserve. Le domaine public maritime de l’État en Polynésie française doit être clairement identifié, réserve faite des éventuelles emprises relevant de la compétence liée à la défense nationale. Il convient aussi de rappeler la compétence de la Polynésie en matière de culture, telle qu’elle résulte de la combinaison des articles 13 et 14 de la loi organique statutaire. Or il semblerait que le dernier alinéa de l’article 2 intervienne dans le domaine de compétence de la Polynésie, puisqu’il vise les biens culturels maritimes dont les éléments sont énoncés par l’article L. 532 1 du code du patrimoine du patrimoine : « Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë. » Toutefois, si une épave ou un vestige pouvant présenter un intérêt préhistorique, archéologique ou historique ne soulève pas de difficultés d’interprétation, il pourrait en être autrement d’un gisement, qui pourrait s’entendre au sens géologique du terme ! À cet égard, pour éviter toute ambiguïté sur l’interprétation de cette disposition ainsi qu’un enchevêtrement des compétences entre

de biens culturels maritimes situés dans son domaine public maritime. Je vous rappelle, mes chers collègues, que cet amendement est soutenu

cette ordonnance est emblématique des difficultés juridiques auxquelles sont confrontées les collectivités d’outre mer et de la difficile appréhension par l’État du droit applicable, souvent peu lisible et accessible. Ainsi, nous devons toujours rester vigilants à l’égard de situations souvent complexes à sécuriser, dans le respect des identités foncières et des évolutions institutionnelles propres à chaque collectivité ultramarine. Pour conclure,

J’ai tendance à le répéter, même si c’est une évidence, car l’attention que nous portons aux situations de nos territoires est singulière et nous caractérise. La Polynésie française est une collectivité d’outre mer régie par l’article 74 de la Constitution. Son statut lui confère une autonomie renforcée et le pouvoir d’édicter des normes relevant du domaine de la loi. Ce statut encadre strictement le domaine d’intervention de l’État, qui conserve des compétences d’attribution limitativement énumérées, tandis que la Polynésie détient la compétence normative de droit commun. Jusqu’en 2019 et depuis le depuis le statut de 2004, l’État disposait d’une compétence normative expresse sur son seul domaine public, et non sur son domaine privé, qui représente pourtant 12,5 kilomètres carrés. Cette répartition des compétences entre territoires et État présentait un caractère inhabituel, au regard des régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre mer. La compétence sur le domaine privé revenait donc, par défaut, aux institutions de la Polynésie, qui n’ont d’ailleurs jamais usé de cette faculté. Comme l’a rappelé M. le rapporteur, dont je salue le travail, la loi organique de 2019 a précisé que l’État était compétent pour fixer les règles relatives à son domaine privé et à celui de ses établissements Le principe de cette extension a, par ailleurs, été approuvé par un avis de l’assemblée de la Polynésie française en date du 15 novembre 2018. pour produire pleinement ses effets juridiques et devenir pleinement applicable, cette réforme impliquait une mise en cohérence globale des dispositions du livre VI de la cinquième partie du code

vis à vis de cette collectivité d’outre mer, qui, certes, a été saisie du projet d’ordonnance, mais dans des conditions compliquées, en plein milieu des élections territoriales. Nous sommes rassurés que notre assemblée ait pleinement joué son rôle et ait pu échanger avec les acteurs locaux, qui ont été écoutés et, surtout, entendus – j’ai été attentif à ce que vient de dire Lana Tetuanui. de l’examen de ce texte pour rappeler l’État à son devoir. Monsieur le ministre, près de soixante ans après les premiers essais nucléaires français dans le Pacifique, les questions des réparations et des compensations pour les dommages causés par ces tests ne sont toujours pas résolues. près de 170 000 personnes ont été exposées à des radiations, les avancées de 2010 ne répondent toujours pas à la triste réalité, sur laquelle j’ai discuté avec plusieurs représentants du territoire polynésien.

Dès 2015, le Sénat a alerté sur cette situation, née du « morcèlement » du droit de la domanialité et d’un « éparpillement des normes applicables dans un grand nombre de textes différents qui interagissent entre eux La Polynésie française n’échappe pas à cette situation. En effet, les compétences de l’État en Polynésie sont régies par le principe d’attribution : la compétence de principe appartient à la Polynésie sur son territoire, tandis que les compétences de l’État lui sont spécifiquement attribuées. La loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française précise, en son article 14, que l’État est compétent pour fixer les règles relatives à son domaine public. Or, comme le précise l’étude d’impact, une lecture stricte de cette disposition pouvait laisser entendre que l’État n’était pas compétent en Polynésie pour fixer les règles relatives à son domaine privé ou au domaine, public ou privé, de ses établissements publics. C’est pourquoi, afin de lever toute difficulté d’interprétation, l’article 3 de la loi organique de 2019 a modifié la loi de 2004 pour conférer explicitement à l’État la compétence relative à ces domaines. Comme le souligne le rapport de la commission des lois, l’assemblée de la Polynésie française, consultée sur le projet de loi organique en 2019, avait émis un avis favorable sur cette évolution. La commission des lois du Sénat jugeait cette clarification de nature à « parfaire la coordination entre l’État et le pays ». L’ordonnance soumise à la ratification du Sénat est la traduction de cette clarification. Les difficultés juridiques auxquelles sont confrontés les outre mer, avec un droit applicable souvent peu lisible et accessible, rendaient cette clarification il faut surtout rappeler que cette clarification ne doit pas empêcher l’adaptation et la prise en compte des spécificités locales et du statut particulier de la collectivité Par ailleurs, la question du domaine public maritime de l’État, soulevée par l’amendement déposé par notre collègue Mme Lana Tetuanui, nous interroge. Le sujet est particulièrement sensible, la Polynésie française étant constituée de 118 îles, réparties en cinq archipels, s’étendant sur une superficie comparable à celle de l’Europe, avec une surface émergée de 4 200 Si la quasi totalité du domaine public maritime en Polynésie appartient à la collectivité et que le domaine public maritime de l’État est très résiduel – quelques installations portuaires affectées à la marine nationale –, il ne faudrait pas que, sous couvert de clarification, ce dernier puisse empiéter sur les compétences de la collectivité. Bravo ! Comment être sûr que l’application de cet article ne présente aucun risque d’intrusion de l’État dans l’exploitation des ressources naturelles présentes dans les sous sols marins Comment en être certain, quand on sait que ces ressources peuvent être considérées comme des matières premières stratégiques et qu’elles pourraient faire l’objet d’une volonté de mainmise de la part de l’État ? Que recouvre exactement la notion de « gisement archéologique », qui est mentionnée mentionnée dans l’ordonnance ? S’agit il, comme nous le dit M. le rapporteur, des seuls gisements au sens du code du patrimoine, c’est à dire constitués « par une épave qui présente un intérêt archéologique » ? Sommes nous sûrs que cela exclut toutes les ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, dont l’exploitation relève bien d’une compétence appartenant à la Polynésie française ? Nous réserverons notre vote aux clarifications qui seront apportées ici sur ce point.

à abroger l’article L. 5621 2 du code général de la propriété des personnes publiques.

organique statutaire, selon lequel « la Polynésie française réglemente et exerce les droits de conservation et de gestion, le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment les éléments des terres rares, des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous sol et des eaux sur jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive ». En effet, au sens géologique, un gisement géologique, un gisement désigne une disposition de couches de minéraux dans le sous sol. Nous sommes entièrement dans la compétence de la Polynésie française ! Tel est le sens de cet amendement. Quel est l’avis

Lors de l’examen du texte en commission, un amendement ayant le même objet a été rejeté, car nous avons estimé que l’ordonnance n’entraînait pas les risques d’empiétement qui viennent d’être évoqués, pour deux raisons essentielles. En premier

mais l’ordonnance précise qu’il n’est applicable à la Polynésie française qu’« en tant qu’il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l’État ». En effet, le code du patrimoine précise déjà que l’acquisition des biens culturels maritimes par l’État ne s’applique en Polynésie française qu’au domaine public maritime de l’État. plus est, le code du patrimoine polynésien prévoit explicitement que la collectivité peut revendiquer des biens culturels maritimes, à l’exception de ceux qui sont situés dans le domaine public maritime de l’État. Enfin, cette compétence donnée à l’État est toute relative, puisque le domaine public maritime de l’État en Polynésie est très résiduel. Il se limite, en réalité, à quelques installations portuaires affectées à la marine nationale.

Un gisement, au sens du code du patrimoine, désigne une épave qui présente un intérêt archéologique, en raison de sa cargaison ou de sa bonne conservation.

pour terminer, que des dispositions identiques s’appliquent à la Nouvelle Calédonie depuis 2016, sans avoir engendré le moindre empiétement.

n’empiète pas non plus sur les compétences que la collectivité détient pour légiférer sur le domaine public maritime qui lui appartient. Bien au contraire, la compétence que détient l’État en métropole est précisément adaptée pour la Polynésie française

de simplifier le droit applicable. Enfin, le code du patrimoine polynésien traite précisément de la question des biens culturels maritimes, notamment de ceux qui sont situés dans le domaine public maritime de l’État, reconnaissant d’une certaine manière l’existence de cette notion.

L’histoire du nucléaire en Polynésie, l’histoire du foncier en Polynésie et, aujourd’hui, l’histoire du domaine public en Polynésie : voilà des sujets qui parlent aux Polynésiens.

le texte de la commission, l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023 389 du 24 mai 2023 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à la Polynésie française. Je rappelle

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est parvenue à l’adoption d’un texte commun.